La séance est reprise. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription de la suite de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance à l'ordre du jour du vendredi 17 mai, le matin, l'après-midi et le soir. Acte est donné de cette demande. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé est parvenue à l'élaboration d'un texte commun.

et une intégration réussie. Il prévoit les différentes façons de satisfaire à l'obligation de scolarité, soit par l'inscription dans un établissement scolaire, soit par le choix d'instruction par la famille, et précise les modalités d'inscription. Son sixième alinéa, issu de la loi susmentionnée, soumet l'inscription de l'enfant à la délivrance d'un certificat par le maire à la famille

constituait pourtant une réécriture intéressante de cette procédure de recours : en cas de refus d'inscription du maire, le Dasen, agissant « sur délégation du préfet », procédait à l'inscription définitive, après avoir requis le maire, comme le prévoit la procédure de droit commun du code présent amendement vise à rétablir ce dispositif en le modifiant légèrement afin de lever une ambiguïté. Il tend ainsi à prévoir que le Dasen pourra apprécier la légitimité du refus du maire sur des motifs explicites et fondés.

211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit la motivation de tout acte administratif restreignant un droit ou l'exercice d'une liberté publique. Nous proposons d'en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale.

Le scrutin est ouvert.

mes interventions centrées sur ma collectivité, mais je pense que vous comprenez la situation très particulière de l'éducation dans ce territoire. Cet article instaure une visite médicale obligatoire pour les enfants de 3 ou 4 ans. C'est important pour repérer divers troubles.

réaliser le bilan par une personne parlant ces langues. Pour autant, ces visites précoces permettraient bien sûr de dépister plus tôt les problèmes de santé, de langage et de communication de nos jeunes élèves, problèmes qui sont bien réels

et modifié en commission au Sénat, vise à instaurer une visite médicale obligatoire à l'école pour les enfants de 3 ou 4 ans. L'intention est louable, sachant que les inégalités de santé sont déjà installées avant l'âge de 6 ans, voire dès

à 4 ans, notamment en école maternelle. Dans ce contexte, il est proposé de ne pas introduire dans la loi une mesure inapplicable et redondante qui constitue une fausse promesse, propre, de surcroît, à rendre illisible le parcours de santé des jeunes enfants. Quel est l'avis de la commission ?

C'est une bonne chose, car ces services sont particulièrement compétents pour la prime enfance, et leur taux de réalisation des visites est bien meilleur que celui des médecins scolaires. Il semble donc de bonne politique de ne pas remettre en cause un dispositif qui fonctionne et a fait ses preuves et de ne pas surcharger inutilement la médecine scolaire. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 405 du Gouvernement.

L'article L. 113-1 du code de l'éducation posait le principe qu'un enfant scolarisé en classe maternelle ou en classe enfantine pouvait, à la demande de ses parents, être scolarisé dans l'école la plus proche de son domicile. le bon sens est parfois galvaudé ... Cet article rappelait à juste titre que le bien-être d'un enfant, quand il a moins de 6 ans, passe aussi par sa scolarisation dans une école située à proximité du domicile, permettant de préserver son temps de sommeil. Or, avec la disparition prévue des classes enfantines, l'exigence de proximité doit être réaffirmée dans la loi.

n'est pas placé dans les mêmes conditions d'apprentissage qu'un jeune urbain, habitant beaucoup plus près de son collège. Ces inégalités se retrouvent en fin de cycle d'apprentissage

pour un aménagement du territoire cohérent et la concrétisation de nos engagements environnementaux issus de la COP21. La sobriété des déplacements doit être une préoccupation de tous les instants dans l'élaboration d'une carte scolaire : moins de déplacements, c'est aussi une facture d'essence et une facture énergétique bien moindres.

Comme le précise l'exposé des motifs de votre projet de loi, monsieur le ministre, « les principes généraux du système éducatif font de l'éducation un droit, de l'instruction une obligation et de l'enseignement un service public gratuit et laïque. Ces principes sont au fondement de notre contrat social et à ce titre sont rappelés dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. » Former les élèves, les futurs citoyens, nécessite des enseignants et, comme le présuppose cet article, des enseignants formés.

Une disposition adoptée en commission prévoit que tout enfant doit pouvoir être accueilli dès l'âge de l'instruction obligatoire dans une école ou un établissement d'enseignement secondaire situé le plus près possible de son domicile. Ce principe pourrait s'avérer très contraignant pour nos collectivités territoriales, qui devront établir une sectorisation scolaire. Par ailleurs, il pourrait remettre en cause des dispositifs visant à renforcer la mixité sociale au sein des établissements Enfin, s'agissant notamment de l'enseignement secondaire, l'établissement le plus proche du domicile d'un élève ne proposera pas nécessairement les enseignements correspondant aux choix d'orientation

contre-productif, non seulement pour l'éducation nationale, mais aussi pour les communes et même pour les familles.

Afin de prévenir les temps de trajet excessifs pour les enfants, dont l'instruction sera désormais obligatoire dès l'âge de 3 ans, et de garantir le maintien des écoles dans les zones les plus isolées, l'amendement a pour objet de limiter le temps de trajet à trente minutes entre le domicile et l'école, soit une heure par jour aller et retour.

En effet, des temps de transport excessifs ne peuvent que nuire à la concentration en classe. Il est nécessaire que le service public de l'enseignement soit présent même dans les zones les plus isolées, afin que tous les enfants aient les mêmes chances de réussite

lecture : « L'instruction obligatoire dans un établissement public d'enseignement doit être possible dans un temps de trajet inférieur à trente minutes entre le domicile de l'enfant et l'établissement public d'enseignement. » Cela

en donner lecture : « L'instruction obligatoire dans un établissement public d'enseignement doit être possible dans un temps de trajet inférieur à trente minutes entre le domicile de l'enfant et l'établissement public d'enseignement.

difficulté à reconnaître un rôle important au directeur d'école. C'est pour moi l'occasion de le dire publiquement et officiellement.

Françoise Laborde. Cet amendement vise à rétablir la mention selon laquelle l'enseignement public dispensé pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit. Pourquoi modifier l'article L. 132-1 du code de l'éducation ? Cette rédaction soulève des interrogations sur la gratuité de l'enseignement dans les établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux, les EPLESF, s'ils venaient à être créés. En effet, la rédaction proposée pour cet article couvre l'enseignement public dans les maternelles et écoles élémentaires, tandis que la rédaction de l'article L. 132-2 couvre les collèges, les lycées et les élèves de classe préparatoire. Cela m'amène au questionnement suivant par quel article seraient couverts les EPLESF ? afin de couvrir l'éventuelle réapparition des EPLESF à l'article 6 . Je ne le souhaite pas, mais il faut bien

du code de l'éducation. Ce dernier prévoit que « l'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré ». L'amendement est donc satisfait par le droit

hier. Chacun peut soupçonner tout le monde de bien des choses ; on peut voir des complots partout. Essayons quand même de croire que les intentions affichées par les uns et par les autres sont réellement les intentions visées. Après, on peut ne pas être d'accord sur les chemins à

que tous les jeunes entre 16 ans et 18 ans auront l'obligation de se trouver dans un cursus scolaire ou de s'inscrire dans une formation professionnelle, que ce soit en apprentissage ou en service civique. C'est une manière de lutter contre le décrochage scolaire, mais aussi de s'assurer qu'à cet âge crucial chacun aura toutes les chances de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Cet âge est crucial, parce que, nous le savons, les jeunes se retrouvent aujourd'hui dans un angle mort de l'action publique qu'il nous fallait réinvestir, alors que nous connaissons chaque année près de 500 000 décrocheurs à l'école. Dans les outre-mer, le service militaire adapté joue un rôle fondamental pour les jeunes connaissant des difficultés, scolaires ou professionnelles, car il intervient précisément à un moment clé de la jeunesse. À cet égard, l'obligation de formation entre 16 ans et 18 ans apparaît comme une mesure résolument sociale, en ce qu'elle favorise l'emploi de tous les jeunes, qu'ils soient diplômés ou non. Nous ne pouvons que nous réjouir de sa présence dans le projet de loi. La parole

la bonne réponse à une préoccupation, qui semble être partagée, de répondre aux enjeux de notre époque. Cette obligation de formation, telle qu'elle est aujourd'hui développée, ne nous semble

Je ne serai pas forcément d'accord avec certains de mes collègues de la majorité, car je soutiendrai cette réforme. Simplement, il faut s'en donner les moyens. Or j'ai en main un communiqué de toutes les missions locales du réseau Île-de-France, qui sont aux abois et ont appelé à plusieurs reprises le préfet de région. connaissent une baisse drastique de près de 45 % du financement de la garantie jeunes et une baisse de 5,5 % de la dotation de fonctionnement,

de compétences professionnelles et d'insertion dans le monde du travail. Un projet d'arrêté de l'administrateur supérieur définissant les modalités précises de mise en place de l'apprentissage à Wallis-et-Futuna devrait être présenté lors de la prochaine session de l'Assemblée territoriale.

solution juridiquement insatisfaisante, qui n'est pas à la hauteur des besoins pérennes de ces élèves, lesquels ont besoin d'un accompagnement professionnalisé et justement rétribué. obligation est aussi problématique en dehors de l'école, car il n'existe aucune aide matérielle pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Je voudrais en quelques mots revenir sur ce qu'a dit Mme Brulin sur l'égarement de la commission. Nous avons travaillé dans de très bonnes conditions. J'en profite pour saluer

: La parole est à M. Stéphane Piednoir. Avant les amendements de M. Grand ou d'autres, il y a un amendement de suppression, qui ne vous aura pas échappé. Monsieur le ministre, j'ai été très attentif à ce que vous avez dit pendant la discussion générale : il faut s'en tenir au texte, et uniquement au texte de cet article,

Cette obligation sera remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement- on comprend -, est apprenti ou stagiaire en formation professionnelle- très bien -, occupe ou recherche un emploi- on vient d'en parler -, effectue un service civique ou se trouve dans un dispositif d'insertion sociale. J'ai posé la question lors de la discussion générale : si l'une de ces cinq conditions n'est pas remplie, où se trouve le jeune ?

Pour dire les choses, ils sont dans la rue ; ils dealent en bas des barres d'immeubles. C'est à cela que l'on veut s'attaquer avec cet article 3.

un certain nombre de jeunes dans des cases qui vont bien. Est-ce qu'avec cela on aura réglé le problème du décrochage scolaire ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'avec cela on s'attaque aux jeunes qui sont dans la rue, et qui font ce que je décrivais ? Évidemment non !

Au départ, j'étais très sceptique face à une obligation faite à des mineurs ; obligation toute relative, puisque dépourvue de sanction.

nous avons compris le sens de cet article et de cette obligation de formation. Certes, il s'agit d'une disposition avant tout symbolique, mais il est parfois nécessaire d'envoyer des signaux forts, particulièrement en direction

est de créer une contrainte collective pour l'ensemble des pouvoirs publics, à savoir l'État sous toutes ses formes et les différentes collectivités qui ont la charge de ces jeunes, afin de coordonner

État, missions locales -pour repérer ces jeunes décrocheurs et apporter des remèdes. Dorénavant, toutes les structures sont capables de formuler des offres. Certains lycées professionnels, par exemple, ont des capacités d'accueil libres pour former à des métiers en tension et peuvent tout à fait proposer des remédiations pertinentes. On a cité aussi les écoles de la deuxième chance. Il y a également tout ce que nous faisons pour l'apprentissage. En somme, bien des perspectives s'offrent

Nous avons voté unanimement cet article ; nous avons même applaudi. Nous savons tous ici, et M. Karam nous l'a dit, qu'aujourd'hui cette disposition n'est applicable en l'état ni en Guyane

dans le régime des objectifs communs, et je suis très fier ici, en tant que parlementaire métropolitain, de pouvoir assigner à l'État des obligations d'accueil des jeunes en Guyane et à Mayotte. Je sais que le président Larcher vient de déclarer : « Ce n'est pas parce qu'on a un cap qu'on a le vent qui amène au cap. » Pour ma part, je trouve qu'il vaut mieux avoir un cap que pas de cap du tout, parce que cela permet d'aller chercher le vent. Tel est l'objectif de cet article.

et de suivi. Il nous paraissait donc opportun, et je sais que nous n'étions pas les seuls, que les CIO participent au contrôle, à l'accompagnement et au suivi des jeunes en situation de décrochage scolaire, mais cet amendement a été « retoqué », ce que nous regrettons. Bref, nous voterons contre l'amendement n°

qui devrait être assuré par les missions locales. Jusqu'à présent, il faut le préciser, ces missions locales n'ont pas de relation de contrainte avec les jeunes qu'elles prennent en charge. Tout repose sur le volontariat et le libre choix. Si les missions locales se voient attribuer la responsabilité d'engagement de ces jeunes, il ne peut en aucun cas leur être assigné un rôle de contrôle ou de sanction. Il ne de responsabiliser les parents dans leur rôle premier éducatif, car les jeunes concernés sont avant tout mineurs, c'est-à-dire sous la responsabilité juridique de leurs parents ou d'un tiers désigné. Les missions locales doivent être centrées sur leur compétence première, qui consiste dans le repérage, la prévention du décrochage des jeunes en difficulté et l'accompagnement le mieux adapté, dotées de moyens clairs et durables. Or, comme cela a déjà été souligné ce soir, le budget global des missions locales pour 2019 est en baisse de 8,25 millions d'euros par rapport à 2018, dans le cadre

que vous souhaitez confier aux missions locales ce rôle de contrôle de la formation des jeunes de 16 ans à 18 ans. Pour avoir accompagné les premières permanences d'aide, d'information et d'orientation des jeunes, pour avoir suivi l'évolution et le vécu des missions locales,

Le scrutin est ouvert.

Lors du débat en commission, durant lequel j'avais déjà présenté cet amendement, j'ai bien entendu l'argument de notre rapporteur. Il estime que, contrairement à la situation des jeunes jusqu'à 16 ans, il s'agit non plus d'instruction obligatoire, mais d'une obligation de formation. Pour ma part, je ne vois pas pourquoi un jeune ne pourrait pas préparer un diplôme en se présentant en candidat libre, par exemple.

à offrir la possibilité à un jeune entre 16 ans et 18 ans de préparer son baccalauréat ou un autre diplôme en candidat libre, en étudiant à domicile en famille ou à l'aide de professeurs particuliers.

le contrôle aux jeunes qui ont dépassé l'âge de 16 ans. Ainsi, un jeune de 17 ans qui prépare le baccalauréat chez lui en candidat libre n'est pas, à proprement parler, instruit en famille.

J'émets donc un avis défavorable, car il est difficile de prendre en compte la notion d'instruction en famille qui n'existe pas au-delà de 16 ans. Attendons de voir comment on pourra résoudre par la voie réglementaire le vrai problème posé par ces trois amendements.

de même nature qu'auparavant. Bien sûr, il y a tout un travail à faire pour amener ces jeunes à la formation. Pour autant, je ne pense pas que l'on puisse considérer que la notion d'instruction en famille s'applique dans ce cas. Après, il peut y avoir des intersections de situations : par exemple, si un jeune suit une formation au CNED et qu'il réside chez ses parents, cela ressemble à de l'instruction en famille et cela correspond aux situations de résolution du problème que nous pouvons souhaiter. Toutefois, ce n'est pas juridiquement de l'instruction en famille.

est à M. le ministre. Par cet amendement, le Gouvernement souhaite revenir à une rédaction simplifiée de l'article 3. Il n'est pas nécessaire d'inscrire dans la loi une liste des établissements ou de catégories d'établissements dans lesquels une scolarisation permettrait de remplir l'obligation de formation. La formulation « établissements d'enseignement public ou privé » permet de couvrir une large gamme de situations de scolarisation. Il s'agit de tous les établissements d'enseignement du second degré ou du supérieur, d'enseignement agricole, de formation à distance ou des unités d'enseignement du médico-social qui accueillent des jeunes en situation de handicap. C'est ensuite par un décret en Conseil d'État que l'on pourra préciser les situations permettant de satisfaire à l'obligation de formation, qu'il s'agisse des situations de formation, d'emploi, d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle ou d'engagement, ainsi que celles dans lesquelles les jeunes pourraient être dispensés

En effet, le critère de recherche d'emploi ne correspond pas à un statut administratif, sauf si le jeune est suivi par un opérateur du service public de l'emploi. C'est justement une situation couverte par la rédaction de l'article, qui précise que le jeune satisfait à l'obligation de formation « lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle ».

d'insertion sociale et professionnelle des cas permettant de considérer que l'obligation de formation professionnelle des jeunes de 16 ans à 18 ans est satisfaite. En effet, le critère de recherche d'emploi peut recouvrir des situations très variées, allant de la recherche active à un affichage sans grand effet pour retrouver réellement un emploi. Par ailleurs, le critère d'inscription dans un dispositif d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou d'insertion sociale et professionnelle permettrait qu'un jeune mineur bénéficiant de la garantie jeunes ou du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie soit considéré comme étant en formation, ce qui ouvre un champ considérable de confusions. Cet amendement permet de simplifier la rédaction de l'alinéa

de nombreux jeunes de 16 ans à 18 ans sont démunis de solution pour retrouver une place dans un établissement scolaire à la suite d'une exclusion définitive, d'un décrochage ou d'une rupture dans leur parcours, voire une maladie. Cette nouvelle obligation sera considérée comme satisfaite notamment si le jeune occupe ou recherche un emploi. Ajouté en commission, le critère de recherche d'emploi risque de vider de sa substance cette nouvelle obligation en permettant au jeune de s'y soustraire très facilement. Je vous propose donc de la supprimer. Quel est l'avis de la commission ?

professionnelle. Or la mention d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle a justement pour objet de prendre en compte les jeunes accompagnés dans l'insertion professionnelle, à l'école de la deuxième chance, dont on peut être membre à partir de 16 ans et non de 18 ans. Il appartiendra au décret d'application de déterminer les dispositifs éligibles. Pour l'ensemble

Il convient de s'assurer que cette nouvelle obligation ne soit pas contournée par la déscolarisation et l'emploi d'un jeune de 16 ans dans l'entreprise familiale, par exemple, pour ne citer que ce cas. Je vous propose de préciser que l'emploi devra inclure une formation qualifiante, ce qui peut s'apparenter à de l'apprentissage, et de bien définir les emplois répondant à cette nouvelle obligation de formation.

L'article 3 nouveau instaure une obligation de formation pour les jeunes de 16 ans à 18 ans- ce qui est louable. Selon l'alinéa 7, le contrôle du respect de l'obligation de formation

cela demanderait une transformation radicale de leurs pratiques. Les auteurs de cet amendement estiment que cette obligation de formation doit incomber soit au service public de l'éducation nationale, car il faut permettre la soit aux conseils régionaux, qui doivent avoir la charge de la formation des jeunes, soit aux conseils départementaux quand il s'agit de mineurs protégés. Cette obligation devrait également être assortie de la mobilisation de financements adéquats dans la durée et la globalité. L'article 3 n'apporte aucune

Monsieur le ministre, dans le cadre de la discussion budgétaire pour 2019, on nous avait annoncé une diminution des subventions attribuées aux missions locales. Nous avons été un certain nombre, sur ces travées, à dénoncer cette

Force est de constater que nous n'avons pas été entendus : les subventions ont diminué de plus de 8,25 millions d'euros. De la même façon, dans le cadre de la loi pour la

Françoise Laborde. Cet amendement a pour objet de prévoir un rappel formel de l'obligation de formation de 16 ans à 18 ans lors de l'entretien effectué avec le jeune décrocheur dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine.

Nous demandons, sans beaucoup d'espoir d'être entendus, compte tenu de la position du Sénat face aux demandes de rapports, que le Parlement puisse être informé, avant 2022, de la façon dont les missions locales parviennent à accomplir leur nouvelle mission de contrôle du respect de l'obligation de formation jusqu'à 18 ans imposée aux jeunes par le présent article. Nous venons de défendre un amendement visant à supprimer cette nouvelle mission imposée par le texte aux missions locales qui, à l'heure actuelle, n'ont déjà pas les moyens d'accomplir leurs tâches. Il nous Il nous semble légitime de demander un bilan de l'accomplissement de cette nouvelle mission et un examen des moyens humains et budgétaires qui auront été prévus pour honorer cette nouvelle compétence. Quel

et même, éventuellement, les partenaires sociaux. Il a vocation à décrire une stratégie partagée sur l'orientation et la formation professionnelles. À ce titre, il peut définir des orientations sur le continuum orientation-accompagnement-formation pour les jeunes les plus en difficulté, qui exigent une attention particulière des pouvoirs publics et des opérateurs qu'ils financent. Dans la mesure où le CPRDFOP embrasse d'ores et déjà tous les publics, les jeunes qui seront soumis à l'obligation de formation, il n'est pas utile de compléter l'article L. 214-13 du code de l'éducation. En outre, l'ajout qui est proposé au 3° du I de cet article se rattache au seul champ de la formation professionnelle initiale, alors que l'obligation de formation que nous envisageons a une

Voilà des jeunes qui sont en décrochage, qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas d'avenir, et on leur dit qu'on va les former. Ils ont échoué dans la formation or tout ce qu'on leur propose, c'est l'obligation d'aller pointer à la mission locale, qui n'aura pas les moyens de les suivre et qui n'aura pas de projet à leur

les classes des établissements privés sous contrat dans les mêmes conditions que les classes correspondantes dans l'enseignement public. La baisse de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans obligera donc les communes à prendre en charge également les classes de maternelle des établissements privés sous contrat, alors qu'elles ne le faisaient jusqu'à présent que pour les écoles élémentaires. Cette mesure risque d'accentuer la fuite des élèves issus des classes socioprofessionnelles favorisées vers le privé dès le plus jeune âge. Elle représente par ailleurs, pour certaines communes, une charge financière importante dans un contexte où nombre d'entre elles déplorent déjà le manque de moyens à leur disposition pour entretenir convenablement les locaux et développer l'accompagnement dans les établissements publics. Cet amendement vise donc à dispenser les communes de cette nouvelle obligation de prise en charge des classes maternelles des établissements privés sous contrat.

maternelles ; seules les dépenses liées aux classes élémentaires des établissements privés sous contrat seraient prises en charge dans les mêmes conditions que les classes correspondantes dans l'enseignement public. Cet amendement tend donc à remettre en cause le principe de parité fixé en 1959 de la commission est donc évidemment défavorable : il ne me semble pas opportun de revenir sur ce principe fondamental.

de nouveau au nom de mon collègue Robert Laufoaulu. Cet article prévoit que l'État compensera le surcoût résultant pour les communes de l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire. À Wallis-et-Futuna, il n'y a pas de communes, mais seulement des circonscriptions. Les aides maternelles sont prises en charge par les circonscriptions, alors même qu'aux termes du statut du territoire résultant de la loi du 29 juillet 1961, l'enseignement est à la charge financière de l'État. Les circonscriptions de Wallis-et-Futuna ne sont déjà pas en mesure d'assurer la gestion des aides maternelles, qui pèse lourdement sur leur budget. Comment feront-elles pour assumer le surcoût ? Comment pourront-elles également assurer la formation de ces personnels, telle qu'elle est prévue à l'article 3 de ce projet de loi ? Monsieur le ministre, les élus comme les autorités coutumières et les chefs des circonscriptions de Wallis-et-Futuna souhaitent que la gestion des aides maternelles soit retirée aux circonscriptions pour être confiée au vice-rectorat.

le présent amendement vise à préciser selon quelles modalités pourra être ajusté dans le temps l'accompagnement financier prévu en faveur des communes qui auront connu une augmentation de leurs dépenses obligatoires en raison de l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Afin de lever toute ambiguïté, nous entendons préciser de nouveau que l'augmentation de ces dépenses obligatoires s'appréciera par rapport aux dépenses obligatoires prises réellement en charge au cours de l'année scolaire 2018-2019. Nous réaffirmons que l'accompagnement par l'État revêt un caractère pérenne. de rendre possible, pendant trois ans, à la demande des communes intéressées, la révision de l'accompagnement par une comparaison entre les dépenses de l'année scolaire 2018-2019 et celles des années scolaires 2019-2020 et, le cas échéant, 2020-2021 et 2021-2022. Ce schéma permettra de répondre à la demande de souplesse et de fluidité dans la gestion des demandes d'accompagnement, sans pour autant instaurer de manière excessivement durable un circuit de réexamen annuel qui serait très lourd pour les communes comme pour les services de l'État. Eu égard à la baisse démographique forte et soutenue dans le premier degré au cours des prochaines années, en réalité, seule une minorité faible et décroissante de communes aura intérêt, en tout état de cause, à activer ce dispositif de révision pluriannuel. repris dans le présent amendement la précision issue des discussions de votre commission : « en tenant compte, pour les collectivités qui y procédaient antérieurement à la présente loi, de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées liées à l'État par contrat. » Cette Cette disposition ne m'apparaît en effet ni nécessaire ni justifiée, puisque le dispositif présenté par le Gouvernement, qui repose sur la comparaison entre dépenses obligatoires réellement effectuées entre les années scolaires 2018-2019 et les années suivantes, intègre nécessairement les dépenses relatives aux maternelles privées sous contrat, ce qui prive cette mention de tout objet. De plus, si l'objectif implicite était d'intégrer dans le calcul de l'accompagnement des dépenses d'ores et déjà obligatoires, c'est-à-dire le forfait communal déjà dû dans sa totalité en cas d'accord donné par la commune au contrat passé entre la maternelle privée et l'État, mais non ou incomplètement acquittées à ce jour, cela contreviendrait à la constitutionnalité même du nouveau dispositif, qui ne peut porter, pour les enseignements public comme privé sous contrat, que sur les dépenses nouvelles rendues obligatoires par l'extension de compétences prévue par la présente loi. Enfin, comme l'a proposé M. le rapporteur, supprimer la disposition législative issue des travaux de l'Assemblée nationale relative au cas de la substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à une commune dans l'exercice de la compétence scolaire. Une telle disposition serait en effet redondante avec d'autres dispositions du code de l'éducation. Ainsi, le présent amendement tend à clarifier encore plus les modalités d'accompagnement financier prévues en faveur des communes dans le cadre de l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire.

exerçant la compétence scolaire les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'ils ont prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire précédente, dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Je crois qu'il faut vraiment nous en tenir au cadre qu'a précisé M. le ministre : l'État compense

Toutefois, les services de cet agent peuvent éventuellement être répartis sur plusieurs classes, en fonction des moyens mis en oeuvre par les municipalités. Les pratiques des communes sont à cet égard assez diversifiées. Du fait de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, des communes pourront être amenées à recruter un ou plusieurs Atsem supplémentaires.

Tout a été dit sur l'amendement de Mme Cartron, qui vise à supprimer la prise en compte des forfaits versés aux écoles privées sous contrat par les communes.

entre des collectivités et l'État. Il ne me paraît pas nécessaire dans la mesure où le ministre s'est engagé à ce que les dépenses supplémentaires liées à l'abaissement à 3 ans de l'âge de l'instruction obligatoire soient exclues des mécanismes de limitation

Mes chers collègues, monsieur le ministre, je vais lever la séance. Nous avons examiné 84 amendements au cours de la journée ; il en reste 250 à examiner. La suite